en raison de la reprise tardive de nos travaux, je vous propose d'ores et déjà d'ouvrir la nuit et de siéger jusqu'à une heure quinze afin d'aller plus avant dans l'examen de ce texte. Il n'y a pas d'observation ? La séance est reprise. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Celle-ci préconise de rétablir, dans le cadre de la réforme du compte personnel de formation, la prise en compte des formations des sapeurs-pompiers volontaires au titre de la formation professionnelle continue prévue par le code du travail. Une telle prise par la dernière réforme de 2014, dont il nous appartient aujourd'hui de lever les obstacles. Cet amendement vise à préciser l'éligibilité des formations des sapeurs-pompiers volontaires au compte personnel de formation en confirmant la possibilité d'un abondement des droits déjà inscrits dans les conditions prévues au II de l'article L. 6323-4. L'amendement

Certaines formations de sapeurs-pompiers volontaires font partie des certifications et habilitations qui sont enregistrées au répertoire spécifique, et donc finançables sur les droits au CPF. Il me semble donc plus sûr de leur ouvrir tout le champ du CPF

faisant l'objet d'une discussion commune ont sensiblement le même objet. La commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 2 rectifié de Mme Troendlé, car il lui est apparu nécessaire de préciser que les formations destinées à permettre aux sapeurs-pompiers volontaires d'exercer leur mission sont éligibles au CPF.

l'éligibilité au compte personnel de formation aux parcours de formation reconnus par les branches professionnelles. Par analogie avec les dispositions prévues pour les demandeurs d'emploi en vertu desquelles sont éligibles au CPF les « formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 », le présent amendement vise à rendre éligibles au CPF, pour les salariés, des parcours de formation reconnus par la commission paritaire nationale de l'emploi de leur branche professionnelle comme permettant d'accompagner leur évolution ou leur promotion professionnelles.

inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. Les certifications de branche sont éligibles au CPF à condition que les partenaires sociaux fassent la démarche de les inscrire audit répertoire. Il s'agit d'inscrire l'utilisation du CPF dans une logique

Même avis défavorable. J'ajoute que c'est la position des partenaires sociaux que vient de rappeler Mme la rapporteur, adoptée dans le cadre du dernier accord national interprofessionnel. Je crois qu'il faut les suivre sur ce sujet.

ou incohérence ? Nous nous interrogeons sur les motifs de la suppression de l'article L. 6323-7 du code du travail, qui garantit la mise en oeuvre du droit à une formation initiale différée pour les jeunes les plus fragiles le CPF.

d'une durée complémentaire de formation qualifiante. Si au cours du précédent quinquennat nous avons réussi à réduire le nombre de jeunes sortant sans diplôme du système scolaire en le faisant passer en dessous de la barre des 100 000, nous ne pouvons aujourd'hui nous priver d'un outil qui offre une seconde chance, une chance différée aux jeunes les moins favorisés dans la vie et les moins armés pour construire leur vie d'adulte. Je rappelle à cet égard une donnée qui est désormais largement reconnue : notre système scolaire fait partie des plus inégalitaires, et le déterminisme social y est très prégnant, 60 % des enfants d'ouvriers n'ont pas le bac contre 13 % chez les enfants de cadres. Donner une seconde chance en assurant le droit au retour en formation initiale pour les décrocheurs participe de la lutte contre ces déterminismes Donner plus de droits à ceux qui en ont le plus besoin devrait être le fil conducteur de cette réforme. La suppression de ce dispositif semble être une preuve que le projet de loi va à rebours de cette exigence. Il n'y a pas que ceux qui osent et qui entreprennent qui doivent pouvoir

il consiste à ajouter des heures au CPF des jeunes sans qualification pour les débiter immédiatement au titre des formations assurées par les régions. d'aucun financement spécifique. Dès lors, sa suppression n'aura aucun impact. Les régions pourront continuer à financer ces formations sans qu'il soit nécessaire de les inscrire au CPF des intéressés. Pour le dire plus simplement, le droit à la formation n'est pas supprimé, mais il n'apparaît pas nécessaire de prévoir que ce droit soit mis en oeuvre par le biais d'un abondement CPF. L'avis est donc défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Même avis,

sur la cohésion sociale et sur le déterminisme social, il faut que nous nous en donnions les moyens. Nous n'y parviendrons pas en supprimant petit à petit, quelles que soient les raisons que vous avancez, les dispositifs qui étaient censés apporter un peu d'amélioration et d'épanouissement à ceux qui en ont le plus besoin.

Mme Maryse Carrère. Nous proposons que les salariés qui le souhaitent puissent disposer de leurs jours de repos pour abonder leur compte personnel de formation par le versement des droits acquis dans leur compte épargne-temps dans une limite de dix jours par an. Cela permettrait d'aider les salariés qui n'auraient acquis pas les droits nécessaires à la réalisation de leur formation.

La commission a donc souhaité connaître l'avis du Gouvernement afin qu'il nous indique comment il compterait mettre en oeuvre cette mesure. Quel est l'avis du Gouvernement ?

en aucun cas de confisquer celui-ci par un accord d'entreprise. En effet, la coconstruction n'implique pas l'abandon du principe du consentement des salariés à l'usage de leur compte personnel de formation. Cet amendement vise donc à préciser, dans le cadre d'une démarche de coconstruction entre l'employeur et le salarié, que le CPF est mobilisé dans le respect des conditions prévues

rappelé, ma chère collègue, il s'agit d'un compte individuel. Cet amendement vise à compléter le dispositif de cofinancement du CPF prévu par les travaux de la commission. Il n'est bien entendu pas question de permettre à l'employeur de contraindre le salarié à mobiliser son CPF contre son gré.

amendement, nous poursuivons un objectif d'incitation à l'abondement par une simplification du circuit financier pour les entreprises. En effet, pour favoriser le développement d'accords d'entreprise et de groupe prévoyant des abondements complémentaires, il est essentiel de permettre une gestion simplifiée de ceux-ci. À ce titre, il convient de prévoir la possibilité pour l'entreprise ou le groupe d'en confier la gestion à son opérateur de compétences, en lien avec la Caisse des dépôts et consignations.

pour lesquelles l'employeur abonde le CPF. En effet, le texte issu des travaux de la commission prévoit que l'employeur qui décide d'abonder le CPF de ses salariés dans le cadre d'un accord prend en charge l'intégralité des fonds et bénéficie d'un remboursement par la Caisse des dépôts et consignations à hauteur des droits inscrits au CPF du salarié. Par cet amendement, l'employeur devrait verser l'abondement à l'opérateur de compétences, qui devrait ensuite demander le complément à la Caisse des dépôts et consignations.

Ainsi, je reprends l'exemple du bilan de compétences indispensable à toute transition ou reconversion professionnelle et qui est très parlant. Aujourd'hui, un bilan de compétences, d'une durée de vingt-quatre heures, demain, il ne pourra l'être qu'en trois ou quatre ans, à raison de 1 500 à 2 600 euros. Les 500 euros annuels annoncés sont loin d'être équivalents aux trente-cinq heures souhaitées par les partenaires sociaux. Ce serait le cas si le coût horaire moyen des formations réalisées dans le cadre du CPF était de 14 euros comme vous l'avez retenu, madame la ministre, mais la réalité l'établit à 37,80 euros, selon les propres documents budgétaires du Gouvernement, pour ce qui concerne les formations prises en charge par les OPCA,

Seconde perte de droits : la revalorisation prévue tous les trois ans. Ces deux éléments cumulés restreignent drastiquement la capacité de formation des salariés le CPF. C'est pourquoi nous préconisons une revalorisation annuelle, afin que les salariés ne soient pas perdants sur tous les tableaux. Car nous sommes désormais dans un monde économique qui évolue à vive allure, sous le coup des innovations technologiques. Dans ce contexte incertain, votre réforme de la formation professionnelle instaure-t-elle un cadre efficient pour s'adapter aux mutations en cours

Magras, pour présenter l'amendement n° 245 rectifié. Le bilan de compétences est une action qui permet au salarié de faire le point sur ses compétences, ses acquis et ses besoins. Il peut donc être utile pour une évolution, y compris au sein de l'entreprise, en vue de contribuer à choisir la formation la plus adaptée aux besoins du salarié. Or, en l'état, si les dispositions du futur article L. 6323-17 du code du travail prévoient de sécuriser la possibilité pour un salarié d'effectuer une formation, tel n'est pas le cas pour les bilans de compétences. Il s'agit donc de viser également les cas de refus de l'employeur si le bilan de compétences doit être effectué sur le temps de travail. Pour certains salariés, en particulier les publics fragiles, le bilan de compétences peut être un facteur déclencheur de la formation, et l'obligation de le réaliser en dehors de son temps de travail peut constituer un frein à cette démarche. Dès lors que l'objectif que vous poursuivez avec ce projet de loi, madame la ministre, est, notamment, d'encourager la mobilité professionnelle, il convient de lever les blocages. La formation et la garantie d'y accéder doivent être considérées comme une globalité : il s'agit de ne pas estimer que seule la première favorise la mobilité professionnelle. Tel est l'objet de cet amendement.

commission a adopté un amendement similaire s'agissant des formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences. Le bilan de compétences étant une action moins longue, il me semble plus facile de l'organiser hors du temps de travail.

Bien que la demande d'absence du salarié ne porte que sur le calendrier, aucune disposition réglementaire ou législative actuelle ne fait mention du nombre de refus d'autorisation.

en cas de refus de l'employeur d'accorder à un salarié une autorisation d'absence pour suivre, pendant le temps de travail, une formation financée dans le cadre du compte personnel de formation. Quel est l'avis de la commission ? Lorsqu'un ? Lorsqu'un salarié souhaite mobiliser son CPF pour suivre une formation sur son temps de travail, il doit demander à son employeur une autorisation d'absence. En effet, si la mobilisation du CPF en dehors du temps de travail est un droit, ce n'est pas le cas lorsque le salarié souhaite s'absenter

on voit mal pourquoi l'employeur serait tenu de motiver sa décision. Je précise que la commission a adopté deux amendements tendant à rendre opposable la demande lorsque le salarié souhaite bénéficier d'une validation des acquis de l'expérience ou d'une formation visant à acquérir le socle de connaissances et de compétences CléA.

la rédaction proposée, l'employeur communique sa réponse à une demande d'autorisation d'absence dans un délai fixé par décret et l'absence de réponse vaut acceptation.

Il s'agit d'un amendement de coordination et de mise en cohérence avec les dispositions relatives aux formations éligibles au compte personnel de formation prévues au I de l'article L. 6323-6 Les termes précis consacrés sont ceux de « formations certifiantes », telles que définies à l'article 4 du projet de loi.

Le texte qui nous a été transmis prévoit que le CPF de transition professionnelle peut être mobilisé pour bénéficier de formations certifiantes, mais aussi, à la différence du CPF classique, de formations qualifiantes ne menant pas à une certification. Il semble donc que le Gouvernement souhaite que les conditions de mobilisation du CPF de transition soient plus larges que celles du CPF. Aussi, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur l'alignement proposé dans cet amendement.

En effet, la volonté du Gouvernement, au travers de la création du CPF de transition professionnelle et de la suppression du CIF, est de simplifier, pour les usagers, l'accès à des formations de qualité, ce qui n'est pas nécessairement le cas des formations qualifiantes, qui ne font pas l'objet d'évaluations quant à leur pertinence au regard de l'objectif de sécurisation des parcours professionnels. Par ailleurs, distinguer plusieurs catégories de formations éligibles, selon que l'on se situe dans le cadre du CPF ou du CPF de transition, serait peu lisible, apporterait de la complexité et porterait atteinte à la cohérence d'ensemble du CPF. Aussi, le Gouvernement est favorable à cet amendement de coordination et de précision. Quel est

Ce dispositif doit alors être proposé au salarié et financé par le CPF de transition professionnelle. Le bilan de compétences est une étape indispensable à toute construction d'un projet de transition professionnelle. C'est pourquoi nous entendons, par cet amendement, sécuriser la démarche au sein du CPF de transition professionnelle. est l'avis de la commission ? Les règles d'éligibilité au CPF de transition doivent être les mêmes que pour le CPF. Il me semble donc que cet amendement est satisfait. Mais il est vrai que la rédaction paraît ambiguë. la commission demande au Gouvernement de confirmer que les bilans de compétences seront bien éligibles au CPF. Si tel n'était pas le cas, elle serait favorable à cette précision.

En revanche, le CPF de transition professionnelle vise non pas à déterminer un projet, mais à le réaliser en vue d'un projet plus long. Dans le cadre du CPF de transition professionnelle, donc d'une reconversion, le bilan doit être effectué avant, et peut alors être opéré dans le cadre du CPF ordinaire, si je puis dire.

n° 259 rectifié . En tenant compte des compétences acquises, la validation des acquis de l'expérience est un levier d'optimisation majeur d'un projet de transition professionnelle. Elle permet au salarié de ne pas être obligé de suivre la totalité du cursus de formation. Cet amendement vise à prendre en considération la validation des acquis de l'expérience et à contribuer ainsi à renforcer la liberté de choix professionnels des salariés.

positionnement préalable favorise la réappropriation par le salarié de son parcours sur la base de ses acquis professionnels. Il permet, en outre, d'ajuster la durée du parcours proposé et de réduire le temps de formation, lorsque cela est possible. Il permet enfin d'optimiser la gestion des ressources financières au profit de l'accompagnement d'autres projets de transition professionnelle. de cet amendement prévoient que le salarié qui souhaite se lancer dans un projet de transition professionnelle bénéficie au préalable d'un positionnement. Je comprends la logique, mais je ne vois pas très bien à quoi renvoie cette notion. De plus, on ne sait pas qui doit assurer ni qui doit financer ce positionnement. Je rappelle que le texte prévoit déjà que le salarié peut bénéficier du conseil en évolution professionnelle. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable.

Pardonnez-moi, mais je n'ai rien compris. Vous vous êtes opposée précédemment à un certain nombre d'amendements visant à favoriser la VAE.

Il convient malgré tout de noter que, depuis les lois de 2014 et 2016, que vous n'avez même pas pris la peine d'évaluer avant de nous présenter votre projet de loi, madame la ministre, le nombre de salariés ou de chômeurs ayant activé un compte personnel de formation a beaucoup augmenté.

en tant qu'intermittent du spectacle, et de statuts d'activité divers tels que ceux de salarié, d'auteur ou d'indépendant. Les partenaires sociaux de la filière ont pris en compte cette spécificité en négociant des accords permettant de compléter les fonds légaux destinés à la reconversion des personnes concernées. J'attire votre attention sur le fait que ces partenaires sociaux ne relèvent pas du champ d'application des accords sur la formation professionnelle conclus à l'échelon interprofessionnel, et qu'ils ne siègent pas au sein des instances paritaires interprofessionnelles régionales.

nous proposons que l'opérateur de compétences agréé, qui dispose d'une expertise en la matière avec la gestion du congé individuel de formation, traite les projets de transition professionnelle. L'amendement

Nous considérons que l'échelon interprofessionnel n'est pas le niveau le plus efficient pour la gestion de l'évolution professionnelle de ces salariés. Il est important que la singularité de notre secteur puisse continuer à s'exprimer dans le domaine de la formation professionnelle.

de transition professionnelle. Je rappelle aussi le rôle essentiel et indispensable que joue l'AFDAS qui, depuis plus de quarante-cinq ans, a su accompagner les salariés permanents et intermittents, ainsi que les entreprises composées majoritairement de TPE, de PME et, plus récemment, d'artistes-auteurs. L'opérateur de compétences doit être en mesure de poursuivre l'accompagnement

Le projet de loi crée des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, qui seront notamment chargées d'examiner les projets de transition professionnelle et d'autoriser leur financement au titre du CPF.

Par ailleurs, je peux comprendre l'argument selon lequel le monde de la culture est très spécifique. Toutefois, si cette spécificité devait justifier la mise en oeuvre de règles dérogatoires pour la prise en charge du CPF de transition, on voit mal ce qui s'opposerait à ce que chaque secteur ou chaque branche

aux secteurs sanitaire, social et médico-social. La plupart des salariés du secteur culturel, qu'ils soient permanents ou intermittents, aspirent le plus souvent

n'a pas été mis en cohérence avec les évolutions apportées par la commission des affaires sociales à l'article 17, à savoir la réintroduction de la taxe d'apprentissage comme composante de la contribution unique, et la suppression de la notion d'aide au développement des formations professionnalisantes. Ainsi, le taux de contribution pour les employeurs de salariés intermittents du spectacle est resté à 2,68 %, comme dans la version initiale du projet de loi, alors qu'il aurait dû être abaissé à 2 du fait de la réintroduction de la taxe d'apprentissage. De même, le taux de 0,08 % a été maintenu au titre du développement des formations professionnalisantes, alors que cette notion a disparu du projet de loi. Il me semble important que le Parlement revienne sur la rédaction de ces dispositions, pour éviter que ces entreprises spécifiques ne soient confrontées à une situation aberrante qui reviendrait, pour elles, à s'acquitter deux fois de la taxe d'apprentissage ! La parole est à Mme

Mme Brigitte Micouleau. Il s'agit d'un amendement de précision. Le salarié qui a changé d'emploi pour inaptitude médicale au travail doit être dispensé de remplir la condition d'ancienneté pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle.

Pour bénéficier d'un financement au titre du CPF de transition, le salarié peut se faire accompagner dans le cadre d'un conseil en évolution professionnelle. Or un bilan de compétences sert précisément aux salariés à définir leur projet.

Cela favorisera de surcroît une bonne articulation entre le diagnostic et la mise en oeuvre d'un projet professionnel. On doit laisser aux salariés la liberté de choisir entre bilan de compétences et conseil en évolution professionnelle pour la présentation de leur projet de transition.

? Le texte prévoit que la personne qui demande à bénéficier d'un projet de transition professionnelle peut profiter d'un accompagnement au titre du conseil en évolution professionnelle. La commission souhaiterait connaître les raisons qui ont poussé le Gouvernement à exclure les bilans de compétences de ce cadre,

? Imposer un délai de deux mois et prévoir que l'absence de réponse vaut acceptation risquerait de conduire la CPIR à être excessivement prudente dans la validation des projets, dans la mesure où, de toute façon, l'acceptation suppose la prise en charge financière. On peut considérer qu'un salarié souhaitant obtenir un congé de formation pour préparer une reconversion professionnelle n'est pas pressé par le temps. Il paraît au contraire nécessaire que son dossier soit examiné avec

instruit les demandes de prise en charge financière et autorise la réalisation et le financement des projets. Lorsque la demande émane d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, nous proposons, par cet amendement, d'associer à cette commission représentant de l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés, l'AGEFIPH, qui a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Il s'agit pour nous d'améliorer la prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées. Quel

la possibilité de choisir l'accompagnement adapté à ses enjeux et à ses besoins. Il ressort de l'étude d'impact du projet de loi que la disparition du congé pour réaliser un bilan de compétences sera compensée par l'éligibilité de celui-ci au CPF de transition.

Il est important de garantir l'égal accès, pour tous les actifs, à un bilan de compétences ou à un accompagnement pour VAE de qualité et d'assurer une mobilisation efficiente des ressources rares sur des actions de formation pertinentes pour les actifs et l'ensemble de l'économie.

pour qui le droit à la formation est aussi synonyme de formalités administratives. Ces dernières seraient dès lors allégées. De même, indépendamment de la situation de l'entreprise, les bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle auraient l'assurance de percevoir normalement leur rémunération.

En effet, le projet de loi prévoit déjà qu'un décret précisera les modalités selon lesquelles la rémunération est versée aux bénéficiaires du CPF de transition, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Ainsi, des dispositions particulières seront déterminées par voie réglementaire pour simplifier et alléger les démarches des petites et moyennes entreprises sans qu'il soit besoin d'en faire mention au niveau législatif. Je rappelle d'ailleurs que le bénéficiaire du CPF de transition professionnelle reste salarié de son entreprise pendant la durée de la formation.

la VAE est un levier de sécurisation des parcours par un moyen alternatif et complémentaire d'accès à la certification professionnelle par rapport à la formation

La commission des affaires sociales a proposé de maintenir les dispositions actuelles, permettant à un employeur d'internaliser la gestion du CPF Nous ne sommes pas favorables à ces dispositions, que nous proposons de supprimer. En effet, l'objectif de la rénovation du compte personnel de formation est d'en faire un outil à la main des personnes, et non des entreprises dans lesquelles les actifs sont employés

mais a été peu utilisé en pratique et a parfois été détourné par certaines entreprises pour ne pas s'acquitter de la contribution à la formation professionnelle continue. Si 8 090 entreprises ont affirmé internaliser la gestion du CPF, seules 58 entreprises entreprises ont réellement été actives, dont 29 caisses autonomes du Crédit Agricole. Le système d'information du CPF géré par la Caisse des dépôts et dépôts et consignations fait état que, au 15 février dernier, seuls 1 056 dossiers de formation ont été saisis par ces entreprises sur les trois années pleines de mise en oeuvre du CPF. Par ailleurs, certains employeurs n'ont, à ce jour, saisi aucun dossier dans le système d'information du CPF. Du point de vue opérationnel, la gestion interne du CPF s'est donc révélée être un dispositif peu efficace pour les entreprises et les salariés. En effet, outre un accord d'entreprise conforme et

permettant de formaliser des dossiers de formation pour les salariés. Surtout, la gestion internalisée rend impossible la mobilisation par le salarié de son CPF de manière autonome : celui-ci est contraint de passer par son employeur, même si la formation est effectuée hors temps de travail.

Cette possibilité s'adresse à des entreprises qui ont une vision claire et structurée des besoins en matière de formation. Compte tenu de la baisse potentielle des droits à la formation qui résulteraient des paramètres envisagés par le Gouvernement pour la monétisation du CPF, la commission a jugé pertinent de la maintenir, au moins à titre

? Le texte prévoit que la Caisse des dépôts et consignations pourra conclure des conventions avec un certain nombre d'acteurs intervenant dans la mise en oeuvre du CPF. L'Assemblée nationale ayant retenu la création de commissions paritaires interprofessionnelles régionales qui auront pour mission

l'avis du Gouvernement ? C'est également un avis favorable. La conclusion de telles conventions permettra de préciser les modalités de gestion et d'articulation entre le système d'information de ces commissions et la Caisse des dépôts et consignations, pour une information fluide et partagée.

En facilitant le versement des salaires et la gestion de la partie administrative, on favoriserait la transition professionnelle et la tranquillité des entreprises. L'article que nous examinons prévoit la création de commissions paritaires interprofessionnelles régionales chargées de valider et d'accompagner les projets de transition professionnelle, d'une part, lorsqu'un actif demande à mobiliser son CPF et, d'autre part, lorsqu'un salarié démissionnaire souhaite bénéficier de l'indemnisation chômage. Il est prévu que les FONGECIF actuels pourront exercer ces missions pendant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2019

collègue. Il s'agit de prendre en compte les démarches individuelles des salariés qui souhaitent prendre en charge eux-mêmes leurs frais

pour les finances publiques, qui plus est en dehors des projets de loi de finances, ne semble pas opportun à la commission. En outre, les réductions d'impôt sur le revenu ne bénéficient par

la formation peut également relever d'une obligation de l'employeur. Par ailleurs, cet amendement a des implications financières qui sont difficiles à évaluer. La commission souhaite donc connaître l'avis du Gouvernement.

Cette possibilité doit permettre aux entreprises, notamment aux TPE et PME, de considérer la formation comme un véritable investissement et non comme une charge. C'est une avancée intéressante.

Construite en vue d'accompagner et d'organiser l'augmentation générale du niveau de qualifications exigée par les mutations du travail, elle renforce encore les inégalités entre les salariés.

on peut noter que, en moyenne, les formations effectuées par des personnes peu ou pas diplômées sont de moindre durée et d'un type plus restreint, par exemple une simple adaptation à un nouvel outil de travail. De fait, la formation professionnelle, vue comme une deuxième chance pour celles et ceux qui n'ont pas poussé loin leur formation initiale, ne remplit pas son rôle. pourquoi le chantier qui s'ouvre doit regrouper un ensemble de mesures allant de la simplification des démarches à la meilleure information, en passant par une mise en disponibilité plus aisée de la part des entreprises, mais il faut aussi aller plus loin pour rattraper un retard aggravé par des années d'inaction. C'est tout le sens de cet amendement, qui vise à favoriser les demandes de départ en formation qualifiante ou diplômante faites par des salariés peu ou pas qualifiés. Cela est d'autant plus important que les inégalités d'accès résultent de la question des qualifications, mais aussi de la taille des entreprises, des types de contrats et de la catégorie socioprofessionnelle des salariés demandeurs. La mesure que nous proposons répond à un enjeu sociétal, celui de la vocation émancipatrice de la formation tout au long de la vie. Elle répond aussi à un enjeu économique, et ce à un double titre. D'une part, je l'ai évoqué, les mutations du monde du travail imposent une augmentation générale du niveau des qualifications ; toute une série de nouveaux métiers émerge continûment et les pratiques évoluent, avec en particulier une importance accrue des métiers d'encadrement. Or le barrage à l'entrée, trop sélectif, prive de nombreux salariés d'un accès à une formation. D'autre part, il est essentiel de rappeler que, en moyenne, plus un salarié

? Je note que cet amendement ne vise que les salariés, ce qui peut sembler curieux. Par ailleurs, la rédaction proposée prévoit un accès prioritaire à la formation, sans préciser comment cette priorité doit se traduire. En outre, l'article L. 122-2 du code de l'éducation satisfait en partie cet amendement, puisqu'il garantit un droit à la poursuite d'études pour les personnes sorties du système scolaire sans avoir obtenu de titre de niveau CAP. La commission

en échange d'activités bénévoles et associatives des salariés, d'accorder des droits à la formation, vous transformez une action altruiste et utile socialement en une formation marchande et intéressée. Au-delà de ces raisons déjà suffisantes pour demander la suppression de l'article 2, nous contestons le choix de la commission des affaires sociales du Sénat de supprimer les dispositions visant à ce que les proches aidants d'une personne en situation de handicap ou en perte d'autonomie bénéficient d'un abondement de leur compte personnel de formation au titre du compte d'engagement citoyen. Ces dispositions, issues d'un amendement de notre collègue Pierre Dharréville, qui a été rapporteur d'une mission parlementaire sur les aidants familiaux, tendaient à inclure, dans les activités bénévoles et de volontariat

quelle branche serait compétente pour déterminer les conditions d'alimentation du CPF et financer les formations des proches aidants. La moitié des aidants ayant eu précédemment une activité professionnelle salariée, cela signifie que toutes les branches concernées devraient négocier sur le sujet et, si nous ne disposons pas actuellement d'un fichier des aidants, le n'est pas possible. En attendant, ce sont surtout des femmes- elles représentent 80 % des aidants familiaux -qui se retrouvent pénalisées en termes de formation, d'évolution de carrière et de reprise d'une activité professionnelle.

La France compte aujourd'hui 11 millions d'aidants, qui interviennent régulièrement auprès d'une personne de leur entourage, dépendante, malade, handicapée ou âgée. Cet engagement leur permet d'acquérir un grand nombre de compétences, qui peuvent leur permettre de se réorienter professionnellement : capacité d'organisation, gestion de l'administration, connaissance du secteur médico-social De fait, il nous paraît important de valoriser cet engagement, au même titre qu'une personne salariée, qui réalise la même activité, bénéficie de droits sur son compte personnel de formation. Tel est l'objet de cet amendement. Le compte d'engagement citoyen semble être le meilleur outil pour valoriser l'engagement bénévole ou volontaire des aidants.

un financeur étatique unique sera chargé de rembourser l'ensemble des droits à la formation financés au titre de ce compte. La disposition sera transcrite en loi de finances pour doter des moyens nécessaires le responsable du programme budgétaire unique qui sera retenu. Ce sera donc plus lisible et plus simple.

Cet amendement vise à supprimer l'obligation de mise à disposition des bulletins de paie sur la plateforme du compte personnel d'activité, le CPA. Après plus d'un an de mise en oeuvre, les consultations par

dans le cadre du compte personnel d'activité. Il me semble que cela constitue une garantie nécessaire pour les salariés qui, pour une raison ou pour une autre, pourraient perdre la trace du bulletin dématérialisé qui leur a été envoyé. Il me paraît donc nécessaire, même si elle est encore peu utilisée, certainement parce qu'elle est

proposé à toute personne souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle et établir un projet d'évolution professionnelle. Il est dispensé par cinq organismes : Pôle emploi, l'APEC, les missions locales, Cap emploi et les OPACIF, qui ont vocation à disparaître dans le cadre de ce projet de loi. L'article 3 a pour ambition de renforcer le CEP. Au vu de l'utilisation réduite de celui-ci et même s'il est monté en charge ces dernières années, ce renforcement est nécessaire. Les deux principales critiques portent sur son déficit de notoriété et son positionnement complexe dans le paysage institutionnel. La réforme proposée présente, à nos yeux, deux points positifs, car elle vise à étendre les missions qui sont confiées au CEP. Tout d'abord, au-delà de la formalisation et de la mise en oeuvre du projet de la personne, le CEP identifiera désormais les compétences de la personne accompagnée.

le SPRO, témoigne de nouveau de la logique de déterritorialisation de la formation professionnelle et d'une recentralisation à l'échelon national, et ce alors même que la formation professionnelle est au coeur des compétences des régions. Pour cette raison, nous soutenons la décision de la commission des affaires sociales de réintégrer le CEP dans le cadre du SPRO. La seconde critique porte sur les appels d'offres que mettra en oeuvre France compétences pour désigner les acteurs privés au plan régional qui pourront être opérateurs du CEP pour pour les salariés. Cette désignation à l'échelon national écarte les régions de ce choix, alors qu'elles sont évidemment à même de connaître les besoins propres à leur territoire. Sur ce point, nous soutenons également la commission des affaires sociales dans sa volonté de laisser aux régions le choix de l'opérateur régional. Enfin, le projet de loi a le mérite de clarifier, à l'article 17, le financement du CEP. C'est une bonne mesure. Toutefois, même s'il n'est pas encore

Au premier abord, cet article a l'air évidemment formidable : garantir à toutes et à tous un droit à l'accompagnement tout au long de la vie. Pour un peu, on se prendrait à rêver d'un service public d'accompagnement des carrières, sauf que, le diable se cachant dans les détails, le texte prévoit surtout une ouverture à la concurrence du conseil en évolution professionnelle jusqu'ici organisé par des structures constituant le service public de l'emploi, au premier rang desquelles l'APEC et les missions locales. L'article 3 ouvre ces prestations aux acteurs privés. C'est finalement assez logique, puisque depuis des années, le budget dédié aux structures assurant le conseil en évolution professionnelle est à la baisse

d'un côté, on assèche le service public et on le fait dérailler ; de l'autre, on commence par rendre possible la présence des acteurs privés jusqu'à ce que ces derniers s'imposent face au service public. Madame la ministre, vous avez dit devant nos collègues de l'Assemblée nationale que votre seul souci était que « le que « le CEP achève de prendre son envol, et qu'un conseil de qualité soit délivré à un maximum d'individus ». Je suis très heureuse de constater que nous partageons une ambition commune.

Certes, on peut discuter de l'appréciation trop souvent restrictive de la notion de mieux-disant, mais le constat montre que le prix est toujours le critère central des appels d'offres ! De fait, la mise en concurrence ne peut qu'entraîner une baisse de la qualité, quand le conseil est fourni dans le cadre d'une course à la rentabilité. Quel

L'article 3 du projet de loi sort le conseil en évolution professionnelle du périmètre du service public régional de l'orientation, et confie de fait son organisation à l'État au travers d'une procédure nationale pilotée par le futur établissement

au moment même où la volonté du Gouvernement est de confier toute l'orientation professionnelle aux régions. Ce choix revient également sur un engagement du 9 février dernier du Premier ministre, qui annonçait la mise en place de cahiers des charges régionaux.

Dans une logique de justice sociale redistributive, le CEP doit être étendu aux personnes en situation de handicap dans le cadre de leur projet de maintien dans l'emploi ou de transition professionnelle.

désinsertion professionnelle et le chômage. La situation de l'emploi des travailleurs handicapés se dégrade régulièrement, avec une augmentation du nombre de chômeurs et une hausse des licenciements pour inaptitude.

que le CEP soit étendu aux personnes en situation de handicap dans le cadre de leur projet de maintien dans l'emploi ou de transition professionnelle. Quel est l'avis de la commission ? Les auteurs ? Les auteurs de ces amendements souhaitent que les personnes en situation de handicap bénéficient du CEP. C'est bien évidemment déjà le cas. La loi prévoit d'ailleurs que les membres du réseau Cap emploi soient des prestataires du CEP, habilités de droit. droit. Ces amendements sont donc satisfaits. De plus, si les personnes handicapées constituent un public prioritaire, il ne me semble pas pertinent de les mentionner explicitement, au risque d'oublier d'autres publics, comme les personnes peu qualifiées. Pour ces raisons, la

Ces agréments ont été fondés sur la capacité de ces opérateurs à accompagner des publics spécifiques de secteurs relevant des organisations reconnues multiprofessionnelles pour ce qui concerne des problématiques liées à ces publics. Depuis plus de trois ans, ces opérateurs ont développé une réelle expertise dans l'accompagnement des salariés de leurs entreprises adhérentes et disposent désormais d'équipes aguerries et d'outils performants pour appuyer les démarches des bénéficiaires de CEP. Afin de tenir compte de ces spécificités, pour que cette capacité d'accompagnement difficilement transférable ne soit pas perdue, et conformément à la volonté affichée par le Gouvernement de renforcer le déploiement du CEP sur l'ensemble du territoire, au plus près des besoins des bénéficiaires, il paraît nécessaire de maintenir les habilitations précédemment délivrées pour bénéficier d'un nombre plus important d'opérateurs du CEP. Par conséquent, il est proposé d'ajouter ces organismes à la liste des institutions, organismes et opérateurs appelés à assurer le CEP.

à assurer le CEP. La commission est au contraire en phase avec le souhait du Gouvernement de contraindre les opérateurs de CEP à dynamiser leurs offres en faisant jouer la concurrence. Il reviendra ainsi à la région de désigner, sur la base d'un cahier des charges national, un opérateur compétent pour l'ensemble des actifs occupés du secteur privé. Par ailleurs, dans la mesure où le CEP doit permettre aux actifs de changer, le cas échéant, de métier ou de secteur, il n'est pas

Au-delà, ils seront appelés à réorienter leur mission d'opérateur de compétences, et je ne doute pas qu'ils sauront mettre à profit les compétences qu'ils ont développées à ce titre. L'avis de

s'agit de reconnaître au réseau des FONGECIF une compétence de droit commun pour délivrer le CEP, au même titre que Pôle emploi, Cap emploi, les missions locales et l'APEC, comme cela était le cas dans le texte actuel sur le CEP,

Sur la forme, les FONGECIF, qui ne sont d'ailleurs pas mentionnés sous cette appellation dans la partie législative du code du travail, n'existeront plus du fait de l'intégration du congé individuel de formation, le CIF, dans le CPF. comme je l'ai dit au sujet de l'amendement précédent, la commission est favorable au resserrement des opérateurs du CEP proposé par le Gouvernement. Je rappelle que les FONGECIF demeureront opérateurs de CEP jusqu'à la fin de l'année 2019 et que leur expertise a ensuite vocation à être reprise par des commissions paritaires interprofessionnelles régionales. L'avis de la commission est donc défavorable. est l'avis du Gouvernement ? Même avis.

M. Martin Lévrier. La montée en gamme de l'accompagnement des salariés dans leurs projets d'évolution professionnelle constitue une priorité nationale. Les partenaires sociaux nationaux interprofessionnels, signataires de l'ANI du 22 février dernier, doivent être impliqués dans la construction du cahier des charges et l'attribution des marchés, au même titre que l'État et les régions. Aussi, France compétences, institution nationale à gouvernance quadripartite, gagne à assumer cette compétence. Le présent amendement vise donc à rétablir la possibilité que, pour chaque région, un opérateur du CEP soit sélectionné par appel d'offres de France compétences. Est ainsi supprimée la mention introduite par la commission des affaires sociales du Sénat tendant à permettre que des opérateurs régionaux soient désignés par le conseil régional, après simple concertation du CREFOP, le

amendement a pour objet de permettre aux OPACIF hors champ de délivrer le conseil en évolution professionnelle durant la période transitoire pour éviter un goulot d'étranglement dans les FONGECIF.

FONGECIF. Cela étant, le Gouvernement souhaite qu'un opérateur régional soit désigné dans chaque région par France compétences. Il a semblé à la commission

économique régional. Les régions ont la compétence « développement économique » et ont déjà beaucoup travaillé sur la formation et l'apprentissage. De plus, si la décentralisation a un sens, il convient de laisser à la région la possibilité de désigner l'opérateur du CEP compétent sur son territoire. Le Gouvernement indique que les régions se sont emparées de la possibilité qui leur était déjà offerte. Néanmoins, la désignation d'un opérateur paraissait moins nécessaire, voire redondante, tant que les FONGECIF étaient des opérateurs de droit. Leur disparition conduira les régions à s'investir davantage pour la désignation d'un tel opérateur.

objet de confier l'exercice du CEP à titre transitoire aux CPIR. Or, si l'opérateur régional prévu par l'article 3 ne sera pas désigné immédiatement, les CPIR ne seront pas non plus en place dès le 1 janvier prochain.

pour les autres salariés. Ces OPACIF sont intégrés dans les OPCA qui recouvrent le champ professionnel concerné. Si le texte actuel du projet de loi prévoit que la mise en oeuvre du CEP peut être assurée de façon transitoire en 2019 par les FONGECIF, devenus commissions paritaires interprofessionnelles régionales, il ne mentionne pas ces structures nationales.

les partenaires sociaux ont souhaité, dans l'accord national interprofessionnel du 22 février 2018, que l'appel d'offres concernant le CEP des salariés soit mené au plan national, tout en prenant en compte les spécificités régionales apportées par les régions, qui sont membres de France Compétences, et ce pour deux raisons.

avec cet article 4, nous sommes de nouveau dans le paradoxe. On sent que le Gouvernement est en plein milieu du gué et ne sait quelle est la rive qu'il veut atteindre. En effet, d'un côté, il annonce vouloir se servir de la formation tout au long de la vie pour sensibiliser les salariés à la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, aux enjeux environnementaux et à l'ensemble des défis sociétaux qui attendent la France, mais, de l'autre, il réduit la formation professionnelle et l'apprentissage à leur conception la plus restrictive. La seule mission qu'il leur assigne, c'est la préparation à occuper un poste. Un emploi, pas un métier, et encore moins une citoyenneté. Comme si le monde du travail ne faisait pas partie de ces lieux où l'on forme des citoyennes et des citoyens ! C'est pourtant la sphère où la plupart d'entre nous passons le plus clair de notre temps. La place du travail est telle qu'aujourd'hui c'est notre emploi qui, par bien des aspects, nous définit et nous situe dans la société. Et cet élément central de notre vie ne devrait pas participer à l'émancipation des citoyennes et des citoyens ... Je trouve cela assez paradoxal. En fait, le Gouvernement ne fait que suivre une dynamique, enclenchée voilà plusieurs années, et qui a vu, petit à petit, la formation professionnelle être réduite au service exclusif de l'employabilité. Aujourd'hui, la formation professionnelle est destinée à permettre l'adaptation à un nouveau poste ou à un nouvel outil de travail, à faciliter la mobilité professionnelle et géographique. Les bilans de compétences et la validation des acquis de l'expérience sont trop souvent unilatéralement unilatéralement au service des besoins de l'entreprise, alors qu'ils devraient davantage prendre en compte les aspirations des salariés. À cet égard, la transformation du congé individuel de formation en compte personnel de formation illustre bien le projet du Gouvernement. Le CIF, avec ses limites, permettait à un salarié ou une salariée de suivre une formation longue, avec maintien de la rémunération et retour en poste ensuite, sur la seule initiative de la personne suivant la formation. Il constituait un outil d'émancipation par sa forme et sur le fond. Or, madame la ministre, vous avez décidé de le supprimer, ne résumant la formation tout au long de la vie qu'à une seule maxime : « par les salariés, pour les besoins des entreprises

J'aimerais revenir plus en détail sur la question de la formation initiale et professionnelle, car c'est un élément marquant du présent article. Celui-ci ne traite de formation initiale que sous le prisme de l'apprentissage, et il me semble qu'ici aussi il y a un écueil. ne partageons pas la théorie selon laquelle il faudrait hiérarchiser les voies d'alternance. L'apprentissage, la formation professionnelle et technologique et la professionnalisation ne répondent pas aux mêmes enjeux. C'est pourquoi leur structuration est totalement différente.

La réforme menée par Xavier Darcos en 2009 l'illustre bien. Alors que 75 % des bacheliers professionnels souhaitent poursuivre leurs études supérieures, il est de plus en plus difficile pour eux de voir leurs souhaits parce que les places dans le supérieur professionnel et technologique sont limitées et qu'elles constituent de plus en plus une option pour des bacheliers généraux désireux de faire un IUT avant d'effectuer une troisième année de licence. Le passage de quatre ans à trois ans de la durée du bac professionnel, en plus des 5 000 suppressions de postes d'enseignants qu'il a entraînées, également les publics les plus vulnérables des lycées professionnels, pour lesquels quatre années étaient et restent nécessaires. Enfin, le contenu même des enseignements a profondément changé, à l'image de l'apprentissage. Le morcellement des compétences professionnelles ramenées à l'exécution de microtâches a fait reculer la vocation de l'enseignement professionnel de former à « penser son métier ». C'est d'ailleurs l'une des causes du nombre important de ruptures de contrats d'apprentissage, les entreprises étant une perte de culture professionnelle. Cet article 4, dans sa conception de la formation tout au long de la vie et de la formation initiale en alternance, accentuera cette régression. C'est pourquoi nous demandons sa suppression.

Il ne me semble donc pas opportun de le supprimer. Par ailleurs, je ne partage pas le point de vue négatif présenté dans l'objet de cet amendement. La commission émet par conséquent un avis défavorable.

Le scrutin est ouvert.

C'est avec constance que je vous présente ce troisième amendement, qui concerne la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Il s'agit de décliner la proposition n° 21 de la mission Volontariat, à laquelle j'ai participé comme coauteur.

les actions destinées aux sapeurs-pompiers volontaires. Il ne me semble pas pertinent d'ajouter une mention aussi spécifique à une catégorie particulière au sein d'un article qui tend, au contraire, à définir de manière générale la notion d'action de développement de compétences.

entrant dans le cadre de la fonction de sapeur-pompier volontaire que celles qui entrent dans le champ d'activité professionnelle principal du sapeur-pompier volontaire. Or ces dernières sont naturellement déjà comprises dans le champ des actions de formation.

Nous essayons, avec le Gouvernement, que nous avons sollicité et alerté sur cette difficulté, d'interpeller la Commission européenne pour que, justement,

continue, sa demande n'est pas reconnue. Mes chers collègues, faites-moi confiance : il est indispensable que ce dispositif soit intégré dans ce projet de loi.

explication de vote. Nous sommes souvent confrontés à des risques naturels majeurs, sur l'ensemble du territoire français et, particulièrement, dans les outre-mer. Les sapeurs-pompiers volontaires jouent un rôle important. C'est pourquoi je suis très favorable

La liste des actions de l'article L. 6313-6 ne comprend pas les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprise, alors que ces actions figurent à l'article

rectifié. Cet amendement vise à rétablir le droit des bénévoles de mouvements coopératifs, associatifs ou mutualistes d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions dans le cadre d'actions de formation.

L'article 4 abroge notamment l'article L. 6313-13 du code du travail qui dispose que les formations destinées à permettre aux bénévoles du mouvement coopératif, associatif, ou mutualiste et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions sont considérées comme des actions de formation. Ces formations seront donc désormais exclues du champ des actions qui entrent dans le périmètre de la formation professionnelle. Aussi, nous proposons de les réintégrer, afin de préserver l'accès de ces personnes à la formation professionnelle et de contribuer ainsi à la professionnalisation et à l'attractivité des structures qui les accueillent.

est définie par un cahier des charges qui fera l'objet d'un arrêté pris par le ministre chargé de la formation professionnelle. Ce dispositif n'est pas nouveau, puisqu'il existe pour le conseil en évolution professionnelle. L'adoption une meilleure articulation des deux dispositifs tout en accentuant la lisibilité des deux prestations.

Depuis le mois de février, il existe en effet un cahier des charges qu'il convient d'entériner par un arrêté. Une telle publication permettra une bonne articulation des deux dispositifs, tout en accentuant la lisibilité de ces prestations. Quel est l'avis de la commission ?